Le donateur, actionnaire ou associé de l'entreprise, peut transmettre à titre gratuit les parts ou actions de l'entreprise qu'il détient aux salariés de l'entreprise grâce au dispositif suivant : dès lors que l'entreprise exerce une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, la donation est consentie à l'ensemble des salariés si ces derniers ont au moins deux années d'ancienneté dans l'entreprise. Le donateur ne peut transmettre plus de 15 % du capital de l'entreprise. Lorsqu'elles ont été acquises à titre onéreux, les parts ou actions mentionnées ci-dessus doivent avoir été détenues depuis plus de deux ans par le donateur ou la société. Les donataires ne peuvent pas détenir plus de 10 % du capital de l'entreprise dont les parts ou actions sont transmises au moment de la réalisation de la donation. Les salariés ont la possibilité de verser les parts

Contrairement au dispositif existant pour les fonds de commerce et les entreprises individuelles, l'exonération n'est pas plafonnée à 300 000 euros. En outre, elle n'est subordonnée à aucune condition de poursuite de l'activité par les repreneurs. Je demande donc le retrait

? Même avis. Pour l'année 2020, le secteur des assurances participe à hauteur de 4 milliards d'euros, selon les comptes du Gouvernement : 400 millions d'euros au titre du fonds de solidarité-

non déductible de l'impôt sur les sociétés avait été appliquée après la crise de 2008 en loi de finances, afin que les assureurs participent au redressement des comptes publics. Elle avait rapporté pratiquement un milliard d'euros à l'époque. Dix ans plus tard, nous escomptons 2 milliards d'euros que nous souhaitons réinvestir

pour garantir des rendements d'argent placé, souvent pendant de longues années, pour donner un complément de revenu au moment de la retraite et garantir une progressivité. Ces placements assurantiels

laisse entendre que, sur la base des déclarations des assureurs, ceux-ci auraient pris des mesures généreuses pour près de 3,5 milliards d'euros. Il conviendra peut-être de consolider le bilan.

est le même que celui que nous avons présenté dans l'amendement n° 4 rectifié, sur la taxation du commerce électronique. Il consiste à observer l'augmentation du résultat d'exploitation pendant l'état d'urgence sanitaire et d'en prélever 80 % par rapport à la moyenne des trois dernières années. C'est pour cela que je dis que ce dispositif est pragmatique

L'Association des maires de France a estimé ces pertes à environ 8 milliards d'euros sur trois ans, dont plus de 5 milliards d'euros dès 2020. Le Gouvernement avait annoncé une aide de 750 millions d'euros.

sur trois ans, et à prévoir une compensation recette par recette- on sait que la globalisation des recettes a pour conséquence qu'un gain sur une recette compense une perte sur une autre. Enfin, il vise, d'une part, à prendre en compte l'impact financier du second confinement et, d'autre part, à compenser les pertes de recettes des EPCI sans fiscalité propre, qui sont exclus du dispositif initial.

à la fois les recettes fiscales et les recettes liées à l'occupation du domaine public. Plutôt qu'un calcul collectivité par collectivité, qui paraissait un peu compliqué, nous avons voté un abattement à hauteur de 21 %, afin de tenir compte des onze semaines de fermeture.

quand ça cogne aussi fort ! Les redevances liées au social, à la culture, au sport et aux loisirs pourraient diminuer de 25 %, soit 2,5 milliards d'euros.

ainsi que les collectivités en bénéficient plus facilement et que les crédits ouverts initialement ne soient pas annulés, comme le souhaite le Gouvernement, et soient bien utilisés en faveur du local. Appuyons-nous sur les collectivités, qui représentent encore plus de 70 % de l'investissement public dans ce pays

Il s'agit d'un amendement de repli, qui vise, sans changer le périmètre de compensation des pertes de recettes, à porter le taux d'abattement de 21 % à 31 %, pour tenir compte de la période de confinement de ce mois de novembre, que l'on ne pouvait pas anticiper en juillet dernier.

l'État se dégrade très fortement, de 135 milliards d'euros, celui de la sécurité sociale de 45 milliards d'euros. Je pense qu'il serait illusoire et démagogique d'expliquer que, des trois acteurs de l'action publique, les collectivités seraient les seules à traverser la crise de manière totalement indemne. Personne ne le croirait, à juste

que le mécanisme soit moins sollicité. C'est plutôt une bonne nouvelle, puisque cela signifie que les recettes fiscales et domaniales des collectivités ont moins baissé que nous ne l'avions craint. De même, comme je l'ai dit dans la discussion générale, les recettes de l'État ont moins baissé que prévu, puisque nous avons intégré un ressaut de fiscalité à hauteur de 2,8 milliards C'est la raison pour laquelle, comme en PLFR 3, le Gouvernement est opposé à l'intégration des recettes tarifaires dans la base de compensation. Nous partageons l'avis du rapporteur général sur l'amendement n° 59. Sans dire

des autorités organisatrices de la mobilité. Nous souhaitons qu'il s'applique dans les mêmes conditions que pour Île-de-France Mobilités, à l'exception peut-être des délais de remboursement, puisque les sommes ne sont

des recettes tarifaires qu'elles tirent de leurs services publics locaux. Le phénomène est particulièrement marqué en ce qui concerne les activités dites « touristiques »- campings, établissements thermaux ... pour lesquelles les pertes de recettes tarifaires sont quasi totales du fait de la fermeture des sites. Les entreprises des secteurs relevant du tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien ou de l'événementiel, qui sont les plus touchées par la crise économique actuelle, bénéficient d'une mesure exceptionnelle d'exonération de cotisations et de contributions sociales. Les régies municipales qui gèrent un service public à caractère industriel et commercial touristique sont exclues de toute mesure de compensation. Au regard de la réduction de leur activité, liée notamment à leur dépendance à l'accueil du public, elles sont pourtant tout autant affectées par les conséquences économiques et financières de la propagation de l'épidémie de covid-19 que les entreprises des secteurs touristiques, hôteliers, etc., cette incohérence se traduit par une dégradation alarmante et durable des finances des communes auxquelles il appartient de gérer ces budgets annexes. cet amendement vise à rendre éligibles au mécanisme de compensation des pertes de recettes tarifaires engendrées par la crise du coronavirus les régies municipales financièrement autonomes et à vocation touristique ou culturelle. Quel l'avis de la commission ? aux pertes de recettes des services de tourisme exercés en régie. La comparaison avec le secteur privé ne me paraît pas pleinement justifiée. En effet, ces services sont gérés par des communes, dont les recettes fiscales ont fait l'objet d'une compensation, alors que le chiffre d'affaires des entreprises, lui, n'a pas été garanti par l'État.

Il me semble néanmoins qu'il convient de traiter ce problème au cas par cas avec les services de l'État, raison pour laquelle, monsieur le ministre, je sollicite votre avis.

Le scrutin est ouvert.

À l'heure où le Gouvernement souhaite accélérer le développement des transports et infrastructures ferroviaires, maritimes ou fluviaux, ainsi que leur transition écologique, il semble indispensable de garantir la pérennité et la sécurité financière de l'Afitf. Cette agence, rappelons-le, contribue au financement non seulement de tous les grands projets d'infrastructures de transport, mais aussi des projets prévus dans la loi de programmation du Grenelle de l'environnement. Son rôle est donc essentiel dans le cadre de la transition vers les mobilités douces et durables et vers le développement prioritaire des transports ferroviaires et fluviaux.

a bénéficié d'une dotation de 250 millions d'euros dans le cadre du PLFR 3 et bénéficie, grâce au présent article 2, de 155 millions d'euros

Les recettes fiscales nettes sont minorées de 52 millions d'euros après l'adoption de l'amendement n° 147 visant à supprimer le reversement au budget général des 52 millions d'euros résultant de la baisse du plafond de l'affectation de TSCA à Action Logement.

relative aux lois de finances et de l'article 47 , alinéa 2, du règlement, lorsque le Sénat n'adopte pas la première partie d'un projet de loi de finances rectificative, l'ensemble du projet de loi est considéré comme rejeté. Personne ne demande la parole ?

hauteur de 300 millions d'euros, des pertes de recettes des établissements recevant du public et des billetteries destinées au secteur de la culture et du sport.

d'agir. Nous le savons toutes et tous, le premier confinement a été terrible pour un certain nombre de femmes. Les violences conjugales ont pris une ampleur encore plus importante. Les suites de ce premier confinement et le second confinement que nous vivons n'ont fait qu'amplifier des situations individuelles devenues insupportables.

dans les propos de notre collègue, je distingue deux choses. Premièrement, il y a effectivement les sommes très importantes que le Gouvernement a mises sur la table en 2020 pour régler le problème de l'hébergement d'urgence en cette période de crise sanitaire. Je pense qu'on peut saluer les efforts fournis, les sommes étant particulièrement considérables.

s'agit de refuser le protocole abusif d'indemnisation de l'entreprise EDF à la suite des fermetures des réacteurs 1 et 2 de la centrale nucléaire de Fessenheim. Un versement de 300 millions d'euros en serait l'une des premières étapes. Ce protocole est abusif, car, en couvrant par cette somme des dépenses de post-exploitation de démantèlement, de reconversion des personnels ou de taxes sur les installations nucléaires de base, nous ferions payer au contribuable une bonne partie des coûts qui auraient dû être supportés par l'exploitant, quelle que soit la date de fermeture. En effet, cet exploitant a déjà normalement provisionné, tout au long des quarante-trois ans d'exploitation, cette somme. Ce protocole est abusif, car il repose sur l'idée fausse d'une fermeture anticipée de deux réacteurs qui seraient plus performants et plus sûrs que jamais. C'est une fiction ! Ces deux réacteurs définitivement arrêtés, respectivement depuis février et juin, étaient en bout de course et ne fonctionnaient, en moyenne, qu'un jour sur trois.

centrales. Les défauts majeurs de Fessenheim demeurent : simple enceinte, piscine de désactivation à l'extérieur, faille sismique, implantation en contrebas du grand canal mitoyen, autant d'éléments qui rendent totalement invraisemblable la fiction fiction d'une indemnisation d'EDF pour un montant de l'ordre de 4 milliards d'euros, comme si ces deux réacteurs avaient pu fonctionner jusqu'en 2041 ! À notre avis, ce protocole est abusif au regard des règles européennes. Ne s'agit-il pas en effet d'un avantage financier important et injustifié à un agent économique, facilitant ses interventions sur le marché de l'électricité et faussant ainsi le jeu de la libre concurrence ? S'engager dans un tel protocole d'indemnisation créerait, pour les finances publiques, un précédent fâcheux dont se réclamerait EDF pour toutes les autres fermetures de réacteurs avant leur cinquante, Merci,

de poursuivre, la crise sanitaire a révélé l'impréparation profonde du Gouvernement, incapable d'assurer la protection des élèves et des personnels, le simple respect d'un protocole sanitaire pourtant insuffisant qu'il a lui-même édicté et, donc, des conditions d'études décentes. Les enseignants comme les élèves ont pourtant déployé un volontarisme à toute épreuve pour assurer une continuité pédagogique. Mais les moyens sont aujourd'hui insuffisants pour assurer des demi-classes, disposer de logiciels et de matériels informatiques adaptés ou même de masques. Dans ce contexte,

D'après les explications que nous avons reçues, les annulations de crédits dans le présent PLFR au titre des dépenses de personnel découlent en fait principalement du recrutement d'agents contractuels en lieu et place d'enseignants statutaires dans l'enseignement agricole et de dépenses

une revalorisation à hauteur de 400 millions d'euros supplémentaires des enseignants du premier et du second degré. Précédemment, M. le ministre nous a également informés de la mobilisation de 25 millions d'euros supplémentaires. Monsieur le ministre,

du monde éducatif

les questions de fraude à l'activité partielle. Nous avons pris certaines dispositions. Le contrôle qui avait été, de fait, supprimé par la réduction à quarante-huit heures du délai d'instruction,

le délégué général de La République En Marche, M. Guerini, affirme que, « pour éviter d'avoir une génération sacrifiée, une prime à l'embauche les concernant est nécessaire, ainsi que l'ouverture du RSA pour les moins de 25 ans ».

Attal : « Ce serait, pour moi, se placer dans un esprit de défaite, pour les jeunes comme pour l'État. Aucun jeune ne grandit avec les minima sociaux comme horizon.

Quand vous donnez une allocation à un chômeur, est-ce que vous lui dites, en le regardant en face : « Je vous donne cette allocation, parce que votre horizon, jeune homme, ou jeune femme, ce sera le chômage toute votre vie » ? Non ! sont privés du droit au travail, on leur donne une allocation, c'est-à-dire un minimum de dignité dans une économie de marché, mais on ne leur dit pas : « C'est votre horizon !

Donnez un horizon à la jeunesse !

inégalités, qui, d'ailleurs, ne sont jamais sources de progrès économique et social ? Il faut absolument répondre, dans l'urgence, à cette situation. C'est bien une réponse d'urgence que nous proposons, une revalorisation de 187 euros par mois, c'est-à-dire supérieure aux 150 euros

et de pertes d'emploi massives. On estime ainsi que, d'ici à cinq ans, la France comptera 1 million de personnes supplémentaires vivant sous le seuil de pauvreté, s'ajoutant ainsi aux 9,8 millions que l'on comptait déjà en 2018. Cette augmentation de la pauvreté s'accompagne d'une hausse importante du nombre d'allocataires du RSA. Dans certains départements, cette hausse dépasse déjà les 10 %. L'éradication de la pauvreté devrait être l'un des objectifs premiers du Gouvernement. Nous proposons donc, par cet amendement, la hausse du RSA au niveau du seuil de pauvreté. cette hausse de 10 % est estimé par l'Observatoire des inégalités à 1,7 milliard d'euros en année pleine, soit 425 millions d'euros par trimestre. C'est un investissement important, mais nécessaire pour permettre la relance dont a besoin l'économie. la commission. Ces trois amendements raisons pour lesquelles j'émets un avis défavorable

est la même que pour les amendements précédents, sur le RSA jeunes : qui paie ? Êtes-vous en train de militer- c'est ce que je comprends -pour une recentralisation du RSA au niveau de l'État qui, lui, agit « quoi qu'il en coûte » ?

certains des prêts garantis par l'État en prêts participatifs afin de lutter contre l'accumulation de ces prêts, qui pèsent de plus en plus lourdement sur les entreprises. Dans un contexte particulièrement difficile pour les entreprises, qui connaissent de nouvelles restrictions dans leur activité professionnelle ou font l'objet d'une fermeture administrative, le risque est que les banques considèrent, à terme, le niveau d'endettement de certaines d'entre elles comme trop important par rapport à leur rentabilité potentielle et n'acceptent plus de signer de nouveaux PGE, malgré la garantie de l'État.

Seraient éligibles à ce dispositif les très petites et petites entreprises qui répondent aux critères cumulatifs suivants : avoir épuisé tous ses moyens d'endettement supplémentaire et se retrouver avec un besoin de restructuration de ses dettes ; faible niveau de trésorerie ; justifier d'une capacité de rebond. Le fonds permettrait aux entreprises de transformer jusqu'à 25 % du montant de leur prêt garanti par l'État en prêt participatif, dans la limite d'un encours total de 40 000 euros. Ce dispositif se distingue des différentes mesures de trésorerie mises en place par le Gouvernement- avances remboursables, prêt garanti par l'État, fonds de solidarité -, car sa finalité L'idée principale, ici, n'est pas d'inonder encore les entreprises de liquidités, mais de commencer à maîtriser leur niveau d'endettement. Cette transformation en quasi-fonds propres aura pour avantage de renforcer la structure de fonds propres des entreprises, de ne pas diluer leur capital de provoquer un effet de levier sur la dette classique, tout en permettant un remboursement sur une longue durée, avec un différé d'amortissement.

Je partage le diagnostic : il faut soutenir les fonds propres de nos entreprises, en particulier de nos PME. Pour autant, je ne suis pas sûr que ce soutien puisse prioritairement par les prêts garantis par l'État. Pourrait remplir ce rôle, en revanche, la garantie que le Gouvernement prévoit d'octroyer à hauteur de 20 milliards d'euros à des fonds investissant en fonds propres

fermés, attendent leur réouverture très prochaine. Cet amendement vise à mettre en place une aide directe au commerçant locataire, au moyen de la création d'un fonds dédié pourvu de 2 milliards d'euros, pour qu'il puisse régler son loyer au bailleur privé.

aux petits commerçants. Cette aide sera versée, à la manière du fonds de solidarité, aux commerces qui ont été fermés administrativement en cette fin d'année 2020 ou qui ont perdu au moins 50 % de leur chiffre d'affaires.

Pour un petit commerçant, le loyer est souvent le poste de dépenses le plus important. Si rien n'est fait, cela pourrait sonner le glas des TPE et PME les plus fragiles. La réponse du Gouvernement ne nous paraît pas suffisante. Certes bienvenu, le crédit d'impôt accordé aux bailleurs repose en effet uniquement sur leur bonne volonté cette mesure simplement incitative nous semble insuffisante pour répondre à cette problématique majeure pour les petites entreprises. Nous proposons donc la création d'un fonds d'intervention pour les loyers commerciaux destiné principalement aux TPE et PME ainsi qu'aux petits bailleurs, ces petits propriétaires, parfois retraités, qui comptent sur les loyers des commerçants. Ce fonds aura pour objectif qu'aucune entreprise ne soit forcée de déclarer faillite en raison de son incapacité à régler son loyer.

Mais, si j'ai bien tout compris- M. le ministre aura certainement l'occasion de le dire -, le Gouvernement, de son côté, propose un crédit d'impôt aux bailleurs.

soit des secteurs considérés comme protégés : hôtels, cafés, restaurants, tourisme, sport, culture, etc. Au-delà de 250 salariés, le crédit d'impôt sera de 50 % également, mais

à 1 milliard d'euros ; il a été intégré par amendement dans le PLF pour 2021, puisqu'il s'agit d'un crédit d'impôt sur une dépense de l'année 2020 qui sera remboursée au bailleur en 2021. Sa place est donc dans le PLF pour 2021 plutôt que dans le PLFR 4. C'est la raison pour laquelle le Gouvernement émet un avis défavorable sur ces deux amendements.

à une solution plus pérenne. J'ai discuté avec quelques présidents de tribunaux de commerce, qui pensent qu'il faudrait instaurer une procédure qui ressemblerait au « rétablissement » tel qu'il existe pour les entreprises individuelles : d'autoriser, sous le contrôle du tribunal et non pas comme dans l'ordonnance du 20 mai 2020, une procédure allégée

aux collectivités locales qui en ont la compétence, plutôt que de toujours vouloir faire, par des impôts nationaux, des choses qu'en définitive vous n'arriverez pas à faire, car les entreprises seront mortes.

Madame Billon,

Sachant que le tourisme représente 30 % du PIB de la Corse, cet amendement vise à créer, une ligne budgétaire nouvelle, un fonds de solidarité abondé à hauteur de 1,5 milliard d'euros à destination des entreprises corses qui dépendent du tourisme. s'agit de soutenir la trésorerie de ces dernières, qui sont particulièrement et dramatiquement impactées par cette crise sanitaire.

ou insuffisances qui sont celles du fonds de solidarité dans un certain nombre de cas. Néanmoins, il me paraît difficile de créer un dispositif spécifique pour une collectivité particulière,

L'ordonnance du 25 mars 2020 a créé un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation. Ce fonds est aujourd'hui un outil permettant de soutenir la trésorerie d'entreprises durement touchées par la crise et qui, sans ce soutien, n'auraient pas pu poursuivre leur activité. Alors que la deuxième vague entraîne de nouvelles restrictions et fermetures, les TPE ont plus que jamais besoin d'un soutien massif et significatif ce fonds de solidarité. dans ce PLFR 4, à un effort massif en prévoyant un élargissement des conditions d'accès au fonds. Cependant, pour beaucoup d'entreprises, le montant de 1 500 euros est insuffisant pour assurer les charges qui sont les leurs, compte tenu notamment du maintien de la condition d'un niveau de perte de chiffre d'affaires de 50 %. Il ne permettra pas de préserver les TPE les plus fragilisées par ce second confinement. L'objet de cet amendement est d'appeler le Gouvernement à accorder des crédits supplémentaires au fonds de solidarité afin que ces 1 500 euros, accessibles aux entreprises qui poursuivent leur activité et qui ne font pas partie des secteurs des listes S1 et S1 , puissent être élevés à 3 000 euros. Par ailleurs, il convient de rappeler que les exonérations de charges proposées dans le cadre du PLFR 4 doivent également concerner les charges sociales personnelles du chef d'entreprise et les charges fiscales de l'entreprise.

prévoir le dispositif le plus approprié possible pour leur permettre de surmonter cette période particulièrement difficile. Dans certains territoires ruraux, il sera très compliqué de se relever de la période que nous traversons.

de l'aide de 1 500 à 10 000 euros pour les entreprises fermées ou celles évoluant dans le secteur très proche et affichant une perte d'activité de 50 %. Cela représente 6 milliards d'euros par mois, soit presque autant que ce qui a été versé aux entreprises pendant toute la période précédente. Cela représentera un

La crise du covid a généré des frais pour les collectivités. Elle engendre également des besoins en termes de moyens informatiques pour éviter les décrochages. Il est donc proposé de créer un fonds à disposition des collectivités locales, sur demande des établissements

Depuis des années, le coût de la vie pour les étudiants augmente plus vite que l'inflation, principalement à cause du prix du logement et des transports. Or les bourses ne suivent pas. Elles ont certes été relevées,

Nous proposons donc une hausse significative des bourses de 10 % pour soutenir les étudiants dans cette période difficile. Concrètement, cela représente une augmentation allant de 10 à 50 euros par mois selon les échelons de la bourse. Un boursier échelon 7 percevrait ainsi 624 euros par mois au lieu de 568 euros actuellement. Cette crise doit nous rappeler à quel point les filets de sécurité sociaux sont essentiels et combien ils ont besoin d'être renforcés. Une augmentation significative des bourses serait un pas important en ce sens.

Villetaneuse explique : « Avant le coronavirus, nous n'organisions qu'une seule distribution par mois. À Paris VIII, on donnait 50 colis maximum. Depuis la première vague, la demande a explosé. On distribue 450 colis toutes les deux semaines aux étudiants de Paris XIII et 1 450 à ceux de Paris VIII. » L'Association fédérative générale des étudiants de Strasbourg, quant à elle, a relancé pour le deuxième confinement les distributions hebdomadaires de nourriture pour les étudiants les plus précaires. première distribution, le 11 novembre, a atteint un record des plus tristes : 1 100 étudiants se sont présentés, soit 400 de plus qu'en mars.

ne pourront pas être mobilisées pour les revaloriser. Je vous propose donc de débattre des montants 2021 alloués aux bourses sur critères sociaux lors de l'examen de la mission « Recherche et enseignement supérieur

survivre durant cette période où ils sont fermés et n'ont pas de chiffre d'affaires. Pour information, au 31 octobre 2020, la baisse de chiffre d'affaires de

du Gouvernement ? Les parcs de loisirs sont éligibles, comme le secteur du tourisme, à l'activité partielle, voire à un taux de 100 % et non de 84 %, puisqu'ils font partie des secteurs protégés, notamment pour les entreprises de moins de cinquante salariés.

De la même manière que M. le rapporteur général a présenté un amendement, que nous avons adopté, tendant à mieux soutenir les toutes petites entreprises et les indépendants,

présent amendement proposent la mise en place d'un fonds d'aide à la quittance. Il permettra d'épauler les locataires les plus fragilisés par la crise et qui ne parviennent plus à payer leurs loyers. L'augmentation prévisible du chômage nécessite des mesures fortes pour empêcher de nombreux Français de basculer dans la précarité. L'urgence aujourd'hui est d'aider les personnes fragilisées par la crise à conserver leur logement. On sait en effet que le logement représente les deux tiers de la consommation préengagée des ménages pauvres. Le « plan de relance » ne signifie pas « sortie de crise », il doit s'accompagner de mesures d'urgence renforcées pour éviter qu'une crise sociale durable ne s'installe. nous proposons un abondement du Fonds de solidarité pour le logement, afin de gérer l'aide d'urgence à la quittance. La gestion de cette aide pourrait être assurée par une cellule d'urgence « crise sanitaire » créée au sein du FSL.

mais un maintien d'une partie de leurs frais fixes. C'est une vraie difficulté, notamment pour les associations et structures d'aide alimentaire, qui sont doublement impactées par la crise dans la mesure où leur public « cible » s'est particulièrement élargi ces derniers mois. mois. Ces associations estiment avoir besoin de 1 milliard d'euros d'aides publiques pour répondre aux demandes auxquelles elles font face sur le terrain au quotidien pour la fin de l'année 2020 et pour 2021. et pour 2021. Nous proposons de provisionner dès cette année la somme de 150 millions d'euros afin que, dans ce contexte si particulier, personne ne souffre de la faim durant le dernier trimestre.

Ils souffrent notamment de charges fixes extrêmement élevées. Il importe donc de leur donner les moyens de faire face à ces charges, car ils sont contraints à la fermeture. Il n'y a pas d'autre alternative que d'avoir recours à des dispositifs spécifiques, puisque les dispositifs généraux ne répondent pas tout à fait à la problématique à laquelle ils sont confrontés.

Cet amendement vise à permettre la mise en place et le financement d'un dispositif particulier de soutien à destination des professionnels des secteurs de la restauration, de l'hôtellerie et de l'événementiel, ces permittents du travail qui exercent dans ces métiers appelés communément les « extras ». Ces salariés qualifiés, issus des écoles hôtelières de France et d'Europe, et qui exercent en contrat à durée déterminée d'usage

l'avis du Gouvernement ?

dit, je suis heureux de la réponse du ministre ; je reviendrai à la charge lors de

Le refus gouvernemental de considérer le livre comme « essentiel » est un acte politique. En effet, le livre n'est pas un objet de consommation comme les autres ; il est un support indissociable de la citoyenneté, un outil d'apprentissage et d'émancipation. Ce refus aura des conséquences concrètes pour les librairies indépendantes, soumises à la concurrence insatiable des grandes plateformes numériques, qui n'offrent pas le même conseil ni le même lien social et qui ne paient pas les mêmes impôts. Ainsi, l'éditeur Denoël évoquait, le vendredi 6 novembre dernier, un chiffre d'affaires des librairies en baisse de 70 % à 85 malgré la procédure de. Cet amendement vise donc à soutenir financièrement les librairies.

payer du personnel pour s'en charger, et le chômage partiel ne leur est que très peu applicable, d'où des coûts supplémentaires. En général, ce sont de petites structures, qui maillent le territoire rural,

ligne et n'ont jamais reculé, y compris lorsque leur tâche nécessitait le contact avec des patients fragiles ou positifs à la covid. Quelque 16 000 salariés ont été exclus de cette prime. C'est une injustice à laquelle il convient de remédier. Quel est

vitrine de la création musicale française à l'étranger ; tout ce secteur culturel est aujourd'hui à l'agonie. Avec l'arrêt des festivals et des établissements de nuit, la vie nocturne comme espace de création est devenue silencieuse.

de Laurent Garnier. Aujourd'hui, se joue la survie de milliers d'artistes et de l'écosystème qui les entoure. Ce secteur pèse plus de 400 millions d'euros. Compte tenu du contexte, ces artistes n'ont pas de perspectives avant très longtemps, et ils passent souvent à travers les mailles des différents soutiens que pourrait leur apporter, notamment, le ministère de la culture.

Gouvernement ? Nous avons déjà dégagé plusieurs centaines de millions d'euros pour le secteur de la culture, et ce PLFR est l'occasion d'octroyer 100 millions d'euros supplémentaires aux industries culturelles. Par ailleurs, la création et les artistes fragilisés font l'objet de dispositions spécifiques dans le cadre du plan de relance. Mme la ministre de la culture

les sujets sont déjà couverts et que nous gagnons à la fongibilité des crédits plutôt qu'à la multiplication de programmes de petite taille, surtout à six semaines de la fin de l'exercice. Cela expliquera mes avis plus lapidaires sur les amendements à venir.

Les producteurs et les fleuristes ont ainsi perdu environ 40 % de leur chiffre d'affaires. Le nouveau confinement tombe au plus mal pour cette filière, car il coïncide avec le deuxième pic d'activité annuelle, qui s'étend de la Toussaint à Noël. Ces pertes sont particulièrement sévères pour les acteurs artisanaux qui n'ont pas opéré leur transition vers le numérique, soit 15 % des fleuristes indépendants, après le premier confinement.

à éviter d'annuler les crédits prévus pour les programmes de recherche et à les redéployer sur le programme « Vie étudiante », pour le financement du plan 60 000 logements étudiants, afin d'accroître le nombre de logements en Crous. Je ne m'étendrai pas sur la situation des étudiants au regard du logement ; nous savons toutes et tous qu'elle est

Cet amendement vise à refuser les annulations d'autorisations d'engagement et de crédits de paiement du programme « Sport » et de les redéployer sur le programme « Jeunesse et vie associative ». Cela permettrait d'augmenter les moyens financiers et humains des associations culturelles et sportives présentes dans les quartiers populaires- politique de la ville -, dont les activités sont d'utilité sociale. Ainsi, le dispositif « Vacances apprenantes », décliné dans le plan Quartiers d'été, dont les actions ont touché près d'un jeune sur trois dans les quartiers prioritaires et qui a été prolongé pour les vacances de la Toussaint, a été apprécié par les communes bénéficiaires. Cela témoigne d'un manque, auquel il s'agit de remédier. Cet amendement tend ainsi à octroyer une dotation supplémentaire à ces communes, qui ont plus de besoins mais moins de ressources. En effet, alors qu'elles disposent de 30 % de capacité financière en moins, leur taux d'imposition est deux fois supérieur et leurs besoins de 30 % supérieurs à ceux des communes similaires ne possédant pas de quartiers prioritaires de la politique de la ville. Cela répondrait

L'augmentation, à 80 %, du taux de prise en charge prévue par le Gouvernement pour les jeunes et pour les habitants de quartiers prioritaires nous semble une bonne chose, mais cela ne répond pas à la situation des associations qui ne sont pas dans ces quartiers et qui font pourtant un travail social aussi important.

nous avons modifié en profondeur les règles d'affectation, aux communes, des recettes de la taxe foncière sur les propriétés bâties. Supprimer une taxe locale et la remplacer par une autre n'est jamais chose aisée, car les différences d'assiette

de l'ancienne taxe d'habitation, en prenant en compte la dynamique des bases imposables. Toutefois, dans le dispositif que nous avons adopté en décembre 2019, le coefficient correcteur ne s'applique pas aux recettes supplémentaires issues d'une hausse des taux communaux

que les communes voteront à partir de 2021. C'est un biais dangereux, qui donne un avantage aux communes ayant des bases importantes grâce à une forte densité économique, au détriment des communes détenant des bases foncières moins importantes et ayant perdu une taxe d'habitation élevée.

Vous le savez tous, ce département a été gravement touché, le 2 octobre dernier, par la tempête Alex, qui a causé des dégâts considérables et qui a sinistré entièrement trois vallées et de très nombreuses communes. Le département des Alpes-Maritimes doit contribuer pour près de 100

le gel de la contribution du département des Alpes-Maritimes au niveau de 2019, soit 64 millions d'euros, et le versement par l'État au fonds d'une compensation de même montant

qu'à hauteur de 120 millions d'euros, alors que, dans le même temps, les DMTO augmentaient de près de 5 milliards d'euros. Nous pouvons tous convenir qu'une plus forte alimentation du fonds aurait certainement été

M. Vincent Segouin. La loi de finances pour 2020 fait de 2017 l'année de référence pour la fixation du montant des transferts de taxe foncière sur les propriétés bâties du département vers les communes à partir de 2021, en compensation de la suppression de la taxe d'habitation. d'habitation. Or, en 2017, à la suite des fusions intercommunales, l'état 1259 a pu faire l'objet d'une présentation inhabituelle, induisant un certain nombre de communes en erreur. Le taux de référence de taxe d'habitation mentionné par l'administration sur cet état s'est fixé à 0 % en raison du retraitement du taux de 2016 par la quote-part du taux de taxe d'habitation départemental transféré dans le cadre de la suppression de la taxe professionnelle. Les communes auraient dû fixer des taux plus importants et percevoir des taxes d'habitation pour 2017. Je rappelle qu'un grand nombre de communes rurales manquent de moyens pour appréhender toute la technicité de la matière. Cette erreur aura des conséquences extrêmement lourdes pour les communes en question- à une petite commune de l'Orne -, puisqu'elles ne bénéficieront d'aucune compensation de la part de taxe d'habitation et devront faire face à la coupe sèche d'une part importante de leurs recettes.

l'avis du Gouvernement ?

il nous paraît indispensable que ces géants du e-commerce contribuent à l'effort national. C'est pourquoi nous proposons qu'ils acquittent en 2021 et 2022 une taxe de 2 % sur leur chiffre d'affaires, afin d'alimenter un fonds de solidarité en faveur des commerces de proximité. Cet amendement ne vise que les entreprises dont le chiffre d'affaires dépasse 25 millions d'euros en France et 750 millions d'euros dans le monde. Les TPE et PME qui choisissent de développer des services de vente en ligne pour compenser la perte des ventes en magasin ne seront bien évidemment pas concernées par cette taxe. L'amendement

distribution. Le groupe Carrefour est en très bonne position, avec une hausse de 3,8 % de son chiffre d'affaires au niveau national et de 8,4 % au niveau mondial au troisième trimestre de

Nous proposons que les acteurs de la grande distribution acquittent en 2021 et 2022 une taxe de 50 % de leurs résultats nets excédentaires par rapport à 2019, afin d'alimenter le fonds de solidarité dont j'ai parlé en faveur des commerces de proximité. Cette mesure nous paraît on ne peut plus raisonnable au vu de la distorsion de concurrence qu'ils Le modèle économique de la grande distribution n'est pas celui du XXI siècle et ne doit pas être celui de l'après-crise. À l'heure où nous devons repenser en profondeur nos modes de consommation et de vie sociale, engageons-nous dès à présent dans un modèle économique plus juste et plus résilient !

fiscales. En Corse, comme dans d'autres zones touristiques, alors que le déconfinement n'a pas permis une véritable reprise, le secteur du tourisme pâtit de nouveau d'un arrêt net de son activité en raison du deuxième confinement. Il faut accentuer l'effort financier à destination de ces secteurs, qui représentent 30 % du PIB de

amendement vise à instaurer une taxe de 10 % sur les réserves de capitalisation des assurances pour les années 2021 et 2022.

l'avis du Gouvernement ?

Il va de soi que, si une entreprise a son siège fiscal ou des filiales dans un paradis fiscal- je veux le dire avec beaucoup de force -, elle ne pourra bénéficier des aides de trésorerie de l'État. » Le

L'avis est défavorable pour deux raisons. Premièrement, le taux choisi ne me paraît pas adapté pour cibler les États et territoires non coopératifs. Le seuil fixé aurait tout de même pour mérite

tant les mesures d'urgence que les mesures de relance sur des bases de justice

Nous ne pouvons pas nous contenter d'aides qui perpétuent un système qui nous mène dans le mur, ni en appeler à la responsabilisation individuelle, qui n'est de toute manière pas suffisante pour résoudre ces enjeux.

l'avis du Gouvernement ?

les amendements que vous proposez sont relativement impraticables, dans la mesure où le recouvrement de la contribution audiovisuelle publique a déjà eu lieu. Par conséquent,

pour intégrer les votes de cette assemblée intervenus lors de cette deuxième partie. C'est l'objet d'un amendement, que le Gouvernement a déposé auprès de votre commission, pendant l'examen a conduit : à ouvrir 25 millions d'euros de crédits de paiement en faveur de la mission « Enseignement scolaire », pour financer le recrutement d'assistants d'éducation supplémentaires dans les collèges et les lycées professionnels ; à minorer à hauteur de 4,7 millions d'euros, les annulations sur la mission « Sport, jeunesse et vie associative et à majorer à hauteur de 500 000 euros les ouvertures sur la mission « Gestion des finances publiques et des ressources humaines ». Par conséquent, le solde budgétaire est dégradé de 30 millions d'euros et se maintient, du fait de l'arrondi, à 224,3 milliards d'euros, comme après l'examen de la première partie. Tel est l'amendement

loi, modifié. En application de l'article 59 du règlement, le scrutin public ordinaire est de droit. Il va y être procédé dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement. Le scrutin est ouvert.